madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat examine ce soir la proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, déposée par le président Gabriel Attal.

L’actualité de ces derniers mois, de ces dernières semaines et de ces derniers jours souligne l’importance de faits graves commis par des mineurs, parfois très jeunes, à l’encontre d’autres mineurs, parfois très jeunes également, et qui suscitent toujours l’indignation et l’incompréhension de tous.

L’État lui même se révèle trop souvent apparemment défaillant, à la fois dans la protection d’une jeunesse en danger et dans la réponse à apporter lorsque cette jeunesse transgresse les règles qui fondent notre société. Nous savons que nous pouvons compter sur l’engagement et le travail remarquables de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne pénale relative à la justice des mineurs : les magistrats, les éducateurs, les greffiers, les avocats, les surveillants pénitentiaires, les acteurs sociaux, ainsi que les policiers et les gendarmes, qui, par leur accompagnement et leur humanité, humanité, s’efforcent de recadrer ceux qui sont nos enfants. Chacun mesure combien notre société est actuellement confrontée à une délinquance des mineurs toujours plus prégnante et à des situations de plus en plus violentes qui heurtent et qui ne sont en aucun cas tolérables.

Ces chiffres se doublent de l’impuissance de l’autorité judiciaire, ainsi perçue par nos concitoyens, qui nous oblige collectivement à réadapter nos méthodes d’intervention et de sanction, sans pour autant renier les objectifs premiers de la justice des mineurs : l’éducation et l’accompagnement. Ne fermons pas les yeux sur les causes de cette délinquance : la précarité, l’isolement et la défaillance de certains parents, les questions migratoires, l’intégration mal réussie, les logements insalubres, les réseaux de prostitution ou de drogue,

Des parents doivent être sanctionnés, parfois parce qu’ils accompagnent même les actes de délinquance de leurs propres enfants, tant certains d’entre eux ont démissionné face à la violence et aux difficultés de la vie.

les entoure. Il s’agit d’éduquer. Des parents sont défaillants, il faut les sanctionner ; des parents crient à l’aide, nous devons les aider. Il nous faut donc réfléchir collectivement à la réponse à apporter, à chaque mesure et à chaque accompagnement mis en place par notre justice à l’encontre des mineurs qui ont besoin de cadre et qui ont surtout besoin que nous les respections. Il nous faut réfléchir collectivement à la façon de renforcer l’autorité, qui va de pair avec l’éducation, une éducation sans sanction ne pouvant que mener aux difficultés que nous connaissons. La délinquance des mineurs est ressentie comme toujours plus forte dans notre débat social, au point d’apparaître comme une tendance inexorable. Gageons que le travail que feront nos deux assemblées permettra à la justice, à l’autorité, de se réaffirmer. Mon prédécesseur, Éric Dupond Moretti, vous a présenté le code de la justice pénale des mineurs (CJPM), qui est entré en vigueur le 30 septembre 2021, avec pour objectif premier de rendre plus lisible et plus cohérent l’ensemble des textes relatifs à l’enfance délinquante.

Il reste beaucoup à faire, mais je salue le travail considérable réalisé par le précédent garde des sceaux et par le Parlement, ainsi que par les magistrats et les éducateurs spécialisés, pour prendre en compte cette demande. La justice pénale La justice pénale des mineurs est régie par trois principes fondamentaux consacrés par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 29 août 2002, et rappelés par l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs que vous avez adopté. Le premier principe est celui de la spécialisation : ce texte ne revient pas, monsieur le rapporteur, sur le principe de la spécialisation des acteurs de la procédure. Les mineurs doivent être jugés par des juridictions spécialisées, selon une procédure appropriée, et c’est une excellente chose. Le deuxième principe est celui de la primauté de l’éducatif sur le répressif, selon lequel un mineur déclaré coupable d’une infraction doit d’abord faire l’objet de mesures éducatives, puis, seulement si les circonstances et sa personnalité l’exigent, de peines.

Les grands principes de rang constitutionnel et conventionnel engagent la France. Quel que soit le gouvernement en place, la France a ratifié et a accompagné la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui a fêté ses 35 ans le 20 novembre dernier. Il s’agit du texte international le plus largement ratifié au monde, par 196 pays, signe de l’importance et de l’universalité des principes Cette convention, notamment son article 40, souligne l’impérieuse nécessité de respecter la spécificité de la situation des mineurs et d’adapter la réponse judiciaire en conséquence.

Dans le cadre de ces travaux sur la réponse pénale à apporter aux mineurs délinquants, un juste équilibre entre ces principes doit donc être trouvé. Tel est l’exercice délicat auquel nous devons nous prêter dans le cadre de l’examen de cette réforme.

Mesdames, messieurs les sénateurs, un mineur délinquant doit être puni. Mais un mineur délinquant est aussi souvent un mineur en danger. Agir sur la délinquance des mineurs implique donc également d’agir en amont au titre de la protection de l’enfance, qui est une politique défaillante des pouvoirs publics.

Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, à une époque où la défiance envers les institutions se fait de plus en plus prégnante, nous devons redonner son autorité à la justice de manière générale, et à celle des mineurs en particulier, tout en garantissant son efficacité sur le terrain et son humanité. La fermeté que nous instaurons est non pas une fin en soi, mais bien la condition indispensable pour restaurer la confiance des citoyens dans notre système judiciaire. Le sujet qui nous réunit aujourd’hui est donc particulièrement sensible. La justice des mineurs ne peut pas être celle des majeurs, mais les mineurs d’aujourd’hui ne sont pas ceux de 1945. Forts de ces deux certitudes, nous saurons trouver de quoi écrire une loi efficace, qui nous permettra un jugement rapide et protecteur.

S’il y a une tendance à la baisse de la délinquance des mineurs ces dernières années, on observe, en revanche, une aggravation préoccupante de la gravité des faits de violence et un rajeunissement de leurs auteurs. Je ne vous donnerai pas de chiffres pour illustrer cette évolution qui voit les mineurs surreprésentés dans les délits ; M. le garde des sceaux vient de le faire. Je ne doute pas, du reste, que chacun d’entre nous a dans sa ville ou dans son département trop d’exemples de cette mutation de la délinquance des mineurs que nous devons nous employer à juguler. Beaucoup d’actions ont été engagées en ce sens. Je pense notamment à l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs,

Je me réjouis, monsieur le garde des sceaux, que vous ayez rappelé les principes de la justice des mineurs. Ces derniers, quand bien même ils dérangeraient certains, sont des principes intangibles :

Dans ce contexte, il n’est pas illégitime que nous examinions un nouveau texte relatif à la justice pénale des mineurs.

La première serait de légiférer sous le coup de l’émotion. Nul ne peut se satisfaire d’une loi édictée à la suite d’un fait divers, impliquant un mineur qui marque l’opinion publique,

serait de mettre de côté les principes constitutionnels spécifiques applicables à la justice des mineurs, dégagés en 2002 par le Conseil constitutionnel et que vous avez rappelés, monsieur le garde des sceaux. Nous n’avons d’autre choix que de composer avec cette réalité. réalité. La proposition de loi votée par l’Assemblée nationale a t elle échappé à ces deux écueils ? La commission des lois a répondu par la négative. Entre les dispositions difficilement applicables et les atteintes aux principes constitutionnels, le compte de la proposition n’y était malheureusement pas. Nous en avons tiré les conséquences en commission, en remaniant certes profondément certains dispositifs et en en supprimant d’autres, mais, parallèlement, nous avons laissé ouvertes de nombreuses initiatives qui seront débattues en séance. Je rappelle à cet égard que nous avons travaillé comme trop souvent dans des délais particulièrement

Le premier volet de la proposition de loi est relatif à la responsabilisation des parents des mineurs délinquants. En la matière, la commission s’est efforcée d’adopter une démarche constructive. Nous avons supprimé la redéfinition des éléments constitutifs du délit de soustraction des parents

nous avons supprimé la sanction civile que le juge aurait pu prononcer à l’encontre des parents ne déférant pas aux convocations qui leur sont adressées en matière d’assistance éducative, notamment parce qu’une telle sanction irait à l’encontre de la logique d’adhésion à la mesure éducative, mais nous avons sécurisé le dispositif en vigueur, en matière pénale. Surtout, c’est le Sénat et le Sénat seul qui a organisé la responsabilité réelle des parents. En faisant participer ces derniers au paiement et au remboursement d’une partie des dommages causés par les infractions, nous avons en effet constitué une véritable responsabilité, sans porter atteinte aux droits des victimes. J’en viens maintenant au second volet de la réponse pénale. Oui, nous avons supprimé la procédure de comparution immédiate telle qu’elle a été adoptée par les députés, considérant que le dispositif ne permet pas d’atteindre l’objectif.

Comme vous le constatez, la commission a donc fait le choix d’expurger ce texte de ses éléments les plus problématiques, afin de repartir sur une base solide – je dirai même juridiquement saine. Oui, les Français attendent

mes chers collègues. Je vous remercie encore, monsieur le garde des sceaux, d’avoir rappelé les principes de la justice des mineurs, qui ne peuvent pas être balayés d’un revers de la main. Je le dis au Sénat Je le dis au Sénat : rien n’est pire que les lois inutiles. Rien n’est pire que les lois inapplicables. Et ceux qui voudraient délibérément ne pas respecter la Constitution, qu’elle est définie par les décisions du Conseil constitutionnel, mettent en cause l’État de droit. Très bien ! La dénonciation facile du gouvernement des juges, qui serait finalement un obstacle à l’action publique, nous amènera demain

Nous avons dans notre code les moyens de lutter. Je le rappelle, les infractions les plus graves relèvent de la cour d’assises et d’une procédure criminelle qui est la même que celle des adultes. En

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter d’un texte qui prétend restaurer l’autorité de la justice face aux mineurs délinquants et à leurs parents. d’une ambition noble et d’un chantier colossal, mais surtout d’un aveu, car, enfin, vous avez compris et vous avez entendu les Français, monsieur le garde des sceaux. L’autorité républicaine s’est évaporée, dissoute au fil des années sous une pluie de laxisme et d’idéologie angélique. Aujourd’hui, que nous proposez vous ? Un texte qui, soyons justes, va un tout petit peu dans le bon sens ; il faudrait être de mauvaise foi pour affirmer le contraire. Responsabiliser les parents, durcir les sanctions, encadrer davantage les mineurs violents. Voilà enfin, peut être, un réveil de la majorité, après des années de sommeil profond. Enfin, la majorité est à l’écoute des Français et de Marine Le Pen. Ce texte ne va toutefois pas assez loin. Il ne fait qu’effleurer la surface d’un problème abyssal : nous sommes face à un immeuble en feu et vous arrivez avec un pistolet à eau, mais surtout avec des années de retard.

parentale. L’assignation à résidence avec bracelet électronique dès 13 ans est peut être la mesure la plus symbolique et la moins contraignante de cette proposition de loi. Un mineur condamné pour trafic de stupéfiants continuera d’organiser son trafic depuis sa chambre,

ce monument d’indulgence en vertu duquel, dans notre pays, un mineur multirécidiviste est encore considéré comme un enfant égaré qu’il faut guider plutôt que sanctionner. Cette ordonnance est désormais trop éloignée des problématiques actuelles.

Vous pensez régler le problème de l’ensauvagement, mais cela n’apporte pas grand chose. Monsieur le garde des sceaux, la France n’en peut plus d’attendre. Pendant que nous débattons, dehors, des citoyens se font agresser, des policiers caillasser et des enseignants insulter en classe.

nous ne pouvons pas commencer l’examen de ce texte sans avoir une pensée pour toutes les victimes, leur famille et leurs proches. Hier soir encore, une rixe en Essonne a emporté un jeune homme de 17 ans. Au nom des membres du groupe Les Indépendants, j’adresse nos condoléances à sa famille. Les violences impliquant des adolescents s’accumulent, transformant des lieux quotidiens en scènes de drame insoutenables. Rixes, agressions, affrontements armés ou trafic ces actes, autrefois exceptionnels, deviennent une réalité trop familière, rappelant l’urgence d’une réponse collective. La justice des mineurs ne saurait être réduite à un débat idéologique. Elle s’impose à nous, portée par l’actualité et par le cri d’alarme des familles, des enseignants, des forces de l’ordre et de la justice. Nous devons mettre en œuvre des solutions. Avant cela, nous devons dresser le constat qui s’impose. La délinquance juvénile est de plus en plus précoce et de plus en plus grave.

Cette réponse, nous la devons à nos concitoyens, car il est de notre responsabilité de les protéger. Mais elle est essentielle aussi pour le mineur concerné, pour le bien duquel il importe de tout mettre en œuvre, afin de tenter d’interrompre la spirale de la délinquance.

L’enjeu est de trouver un moyen de réintroduire davantage de coercition, sans toutefois porter atteinte à nos règles constitutionnelles. Le texte que nous examinons aujourd’hui ne nie pas la dimension éducative, qui doit rester centrale dans notre justice des mineurs.

Ce texte comporte des avancées majeures, que nous soutenons avec détermination. En commission des lois, le travail du rapporteur a permis de préciser et de sécuriser sa rédaction. Nous souhaitons tous ici préserver nos enfants de la délinquance. Pour cela, il faut tout d’abord replacer l’autorité parentale au cœur du dispositif. Lorsqu’un enfant tombe dans la délinquance, ses parents ne peuvent se dérober à leurs responsabilités. à l’encontre des parents si ces derniers négligent volontairement leurs devoirs, notamment en cas de circonstances aggravantes comme la non présentation de l’enfant ou le non respect de l’obligation scolaire. De même, notre groupe soutient pleinement les dispositions du texte visant à mieux indemniser les victimes, sans toutefois exonérer les parents de leurs responsabilités. La réparation des dommages commis par les mineurs n’ayant pas fait l’objet d’un placement incombe en effet à eux de réparer le préjudice aux victimes, ce dont, bien souvent, les assureurs se chargent. Pour ne pas laisser prospérer un sentiment d’irresponsabilité, nous sommes favorables à ce que les assureurs puissent demander aux parents, eux mêmes condamnés pour s’être soustraits à leurs obligations, un remboursement pouvant aller jusqu’à 7 500 euros. Par ailleurs, M. le rapporteur a proposé d’inclure dans le texte plusieurs dispositions concernant les mineurs ayant commis des actes de terrorisme ou de criminalité organisée. Ces mesures nous paraissent nécessaires. Conscients de la clémence de notre système judiciaire à l’égard des mineurs, les réseaux criminels n’hésitent pas à les utiliser de manière abusive. Quand un adolescent de 15 ans est recruté comme tueur à gages, où est notre responsabilité ? Nous devons arracher ces jeunes à l’emprise de ces organisations. Il faut toutefois admettre que certains jeunes, notamment les plus influençables, présentent un profil dangereux. En ce qui les concerne, nous n’avons pas d’autre choix que d’étendre les possibilités de placement, d’assignation à résidence ou encore, le cas échéant, Il s’agit non pas de stigmatiser, mais de reconnaître une évidence : les mesures éducatives ne sont pas toujours efficaces et restent souvent insuffisantes. Il nous appartient de donner à la justice tous les moyens de répondre de manière ferme et responsable. Ce texte n’est pas une remise en cause des principes fondamentaux de notre justice des mineurs. Il ne s’agit ni de traiter les adolescents comme des adultes ni de nier la nécessité d’une approche éducative. Nous devons faire évoluer notre réponse en fonction de la réalité. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de l’adoption de ce texte, pour renforcer les moyens de la justice et mieux protéger notre jeunesse.

Ce texte est bien perfectible, personne ne le conteste. Il constitue cependant un amorçage nécessaire pour lutter contre le fléau de la délinquance juvénile, qui gangrène peu à peu notre pays. Il ne se passe en effet pas un jour sans que les médias s’en fassent le tragique écho. Désormais, c’est très clair, notre indulgence devient notre faiblesse et notre bienveillance se retourne contre nous. Mes chers collègues, à l’évidence, le temps est venu de cesser d’opposer répression et éducation, comme le fait traditionnellement notre système judiciaire. judiciaire. Une sanction immédiate, adaptée et proportionnée revêt nécessairement et intrinsèquement une vertu éducative. Ainsi, il faut sanctionner le mineur le plus tôt possible dans son parcours de délinquance, dès lors qu’il commet des faits répréhensibles, d’une particulière gravité.

Ayons clairement à l’esprit que, désormais, il y a en chacun de nous au moins potentiellement un parent, certes à responsabiliser, mais aussi à rassurer face à une évolution sociétale, hélas ! bien plus rapide que celle de notre politique pénale. Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe Les Républicains voteront en faveur de ce texte. Nécessairement amendé,

sommes ici présents pour discuter d’une proposition de loi sérieuse, qui trouve en partie son origine dans une cause grave : les émeutes urbaines survenues au début de l’été 2023, à la suite du décès de Nahel à Nanterre. L’objectif affiché était double : mettre les parents défaillants devant leurs responsabilités et renforcer l’arsenal répressif dans les situations les plus graves. Sans remettre en cause l’architecture du code de justice pénale des mineurs, réformé en 2021, ce texte redonne un sens aux notions de famille,

d’une mesure équilibrée et responsable, conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2007, laquelle apporte une réponse nécessaire à l’escalade inquiétante de la violence juvénile.

Nous réaffirmons également aux parents qu’ils ne sont pas seuls. La justice n’est pas un ennemi : c’est un cadre qui garantit une réhabilitation sociale à qui veut bien faire cette lecture de son nous tenons à saluer l’engagement exemplaire du personnel de la protection judiciaire de la jeunesse aux côtés de ces jeunes en difficulté. Ses agents contribuent également à faire de la justice des mineurs un levier de réinsertion, tout en prévenant la récidive.

La violence et l’âge sont deux paramètres qui défient notre compréhension de la délinquance juvénile ; l’actualité nous alerte régulièrement sur cette réalité. Or, une fois n’est pas coutume, nous voudrions pouvoir répondre par une nouvelle loi.

Ils situaient la délinquance des mineurs à la croisée de plusieurs politiques publiques, telles que la lutte contre les violences intrafamiliales, l’éducation nationale, la lutte contre la pauvreté, ou encore la politique de la ville. Telle n’est pas du tout l’approche du texte qui a été transmis au Sénat. Cette proposition de loi a un angle, et un seul : la répression. Le député qui en est l’auteur l’affirme d’ailleurs clairement dans son exposé des motifs : « Il nous faut adapter la réponse de notre justice pour provoquer un sursaut d’autorité et une prise de conscience » chez cette partie de nos adolescents qui « glisse […] vers une forme de violence déchaînée, décomplexée, sans règle ». C’est donc sous l’unique prisme de l’efficacité répressive qu’il nous appartient d’étudier ce texte. Notre rapporteur n’a pas manqué de le faire. Ne cédant pas aux sirènes de la communication politique, Francis Szpiner a réalisé un travail de juriste. Il en a tiré des conclusions implacables, que nous ne pouvons que rejoindre – elles vont d’ailleurs dans le sens des amendements que le groupe du RDSE avait déposés en commission –, et qui ont déjà été détaillées. Il a ainsi, notamment, supprimé la comparution immédiate prévue à l’article 4, laquelle n’est pas adaptée à la justice des mineurs et ne correspond d’ailleurs pas à l’architecture du nouveau code

Il ne nous paraît ni souhaitable ni opportun de faire croire aux Français que nous allons avancer grâce à des mesures inadaptées à la réalité de la justice pénale des mineurs. Cette dernière et les pratiques en ce domaine ont d’ailleurs déjà été profondément remaniées récemment, par l’adoption d’un code spécifique entré en vigueur voilà à peine quatre L’évaluation de cette réforme reste à parfaire, et nous regrettons vivement l’absence d’une étude d’impact qui aurait pu nous éclairer. Le nouveau code conserve les principes qui ont guidé notre action en la matière depuis l’ordonnance de 1945 et auxquels mon groupe est profondément attaché. Quels sont ces principes ? Ne pas considérer ni condamner un mineur comme un adulte, car il ne s’est pas encore développé comme tel et n’a pas encore le même sens des responsabilités ; toujours faire primer l’éducatif sur le répressif ; offrir au mineur une juridiction spéciale, avec des juges qui s’attacheront à tenter de l’assagir et à l’insérer correctement dans la société.

toutefois pas tout à fait convaincus de la pertinence de cette vision de l’autorité parentale. Chercher à responsabiliser davantage les parents des mineurs délinquants, c’est omettre le caractère complexe, multifactoriel, de cette délinquance.

Nous croyons également qu’il est illusoire de penser que nous pourrons faire face à ce problème sans nous doter de moyens pour mettre en œuvre les dispositifs qui existent déjà. Tous les professionnels de l’enfance le disent : au pénal comme au civil, nombre de mesures éducatives ou de protection ne peuvent être mises en œuvre faute de moyens.

certains jeunes n’hésitent plus à sortir un couteau pour régler un simple différend. Nous assistons à une véritable banalisation de l’ultraviolence. Rappelons le, 21 % des affaires concernant des mineurs ont pour fondement des faits de coups et blessures volontaires : cette proportion est plus élevée que pour les adultes que nous inquiéter, comme bon nombre de Français, et ce changement de paradigme doit trouver un écho plus fort dans la prise en charge des mineurs par la justice. C’est pourquoi ce texte visait à instaurer, entre autres, une comparution immédiate des mineurs pour les cas les plus graves et à donner plus de facilité aux magistrats pour lever l’excuse de minorité. Toutefois, se pose également la question de la responsabilité des parents dans ce développement de la violence. Bien entendu, nous pensons tous au cas de la mère isolée qui peine à joindre les deux bouts et qui, travaillant de nuit, ne peut pleinement surveiller ses enfants. Dans ce cas, il est impératif que nous n’aggravions pas son fardeau par des dispositions punitives. il faut le dire, certains parents sont démissionnaires et ne s’intéressent ni à l’éducation ni aux fréquentations de leurs enfants. Or l’éducation des enfants relève de la sphère familiale, et il est important de se donner des outils pour le rappeler aux parents.

Pourtant, notre rapporteur a su améliorer certains aspects du texte : je pense particulièrement à l’article 3, qui donne aux assureurs la possibilité de faire participer les deux parents à la réparation financière

souhaitons ainsi rétablir en partie la rédaction de l’article 1, tout en gardant les ajouts du rapporteur, à savoir la suppression de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général, ainsi que l’extension du périmètre de l’actuelle circonstance

l’article 3, si nous souscrivons pleinement au dispositif proposé par M. le rapporteur, nous proposons toutefois une modification. En effet, même quand la mère n’est pas séparée du père, bien souvent le contrat d’assurance est à son nom, surtout s’il s’agit d’une assurance scolaire. Dans la rédaction actuelle, elle serait la seule responsable devant cette assurance. Notre amendement a pour objet que l’indemnisation soit due par les deux parents, quel que soit le signataire du contrat. C’est une mesure d’équité et de responsabilisation de tous les parents. Nous avons également fait le choix de proposer de rétablir les dispositions relatives à la comparution immédiate des mineurs et à l’excuse de minorité. Ce sont les mesures les plus emblématiques de ce texte. Si elles constituent un indéniable durcissement pénal,

de comparution immédiate, que nous vous proposerons également de réintroduire, mes chers collègues, si la césure pénale doit rester la norme, afin de laisser une pleine place aux mesures éducatives, il est nécessaire de sanctionner rapidement les cas les plus graves et de ne pas laisser en liberté, ou du moins sans contraintes, des individus dangereux, quel que soit leur âge. leur âge. Ce texte n’est pas parfait, notamment parce qu’il ne répond pas à la question des moyens, en particulier, monsieur le garde des sceaux, pour la protection judiciaire de la jeunesse, dont les acteurs sont pourtant très engagés et savent faire des merveilles avec des bouts de ficelle. ce texte n’est pas parfait, il n’en est pas moins nécessaire, malheureusement. Face à une délinquance qui évolue plus vite que notre procédure parlementaire et que les procédures judiciaires, il est indispensable que notre justice ne prenne pas plus de retard.

Alors que la société sortait d’une période ultraviolente et particulièrement meurtrière, celle de la Seconde Guerre mondiale, nos gouvernants savaient l’importance de protéger notre jeunesse pour mieux préparer l’avenir. L’ordonnance organisait ainsi la justice pénale des mineurs selon des principes indispensables : l’atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l’âge, la primauté de l’éducatif sur le répressif et la spécialisation des juridictions.

En effet, mettre en cause systématiquement la responsabilité des parents en supposant qu’ils sont forcément démissionnaires, ou même indifférents à l’égard de leurs enfants, ce qui est faux,… Pas toujours ! … est contre productif. Notre groupe luttera toujours contre les parents maltraitants, qui se soustraient à leurs obligations parentales et compromettent la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de leurs enfants. La loi prévoit d’ailleurs déjà de sanctionner ces comportements. Toutefois, les parents de mineurs délinquants ne sont pas systématiquement des parents maltraitants. Les spécialistes du secteur en témoignent : nombre d’entre eux sont contraints parfois de cumuler plusieurs emplois aux horaires décalés, ce qui les empêche, de fait, d’être présents auprès de leurs enfants. Les familles monoparentales sont particulièrement exposées, ce qui ne veut évidemment pas dire que toutes les familles en difficulté ont des enfants délinquants. Ces familles ont avant tout besoin d’un accompagnement social, éducatif, psychologique et juridique. Précisément, que fait l’État pour pallier ses carences ? Cette année encore,

été amputés de 52 millions d’euros cette année. La Cour des comptes alerte pourtant dans son rapport annuel, qui a été publié la semaine dernière, sur les grandes inégalités qui existent dans les politiques publiques à destination de la jeunesse, exposant les enfants au cercle vicieux de la précarité. Cette proposition de loi prévoyait, dans sa version initiale, la mise en place d’une comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans. Outre qu’elle porterait, si elle était adoptée, une atteinte disproportionnée au principe fondamental reconnu par les lois de la République de spécificité la justice pénale des mineurs, cette mesure serait, là encore, contre productive. Elle n’est en effet pas adaptée au temps de l’enfant. Elle ne laisse pas place à la réflexion et empêche toute possibilité pour l’enfant de changer grâce à un accompagnement.

On interdit aux personnes de moins de 16 ans de voter, mais on considère qu’elles peuvent être jugées comme des adultes… Comment le comprendre ? Cette surenchère nous paraît vaine. Monsieur le rapporteur, nous souscrivons à vos constats et nous saluons votre lucidité sur ce texte. Les amendements que vous avez fait adopter en commission ont permis d’éviter le pire, et nous nous en réjouissons. Nous restons toutefois opposés à l’article 4 , qui assimile les enfants de moins de 16 ans à des majeurs lorsque l’infraction est grave. Un enfant de 13 ans ne peut pas être considéré comme un adulte

S’il nous semble par conséquent inévitable en l’état de voter contre ce texte, nous resterons très attentifs à l’évolution des débats, afin qu’aucune modification substantielle particulièrement problématique ne soit votée. La parole

Le Conseil constitutionnel fera son office, mais la politique, ce n’est pas être juriste avant les juristes. » Je pense au contraire que le politique, quand il est législateur, doit faire attention au droit, à sa bonne rédaction et à ses conséquences.

encore une pure mesure d’affichage, de posture de force, de réponse dans l’immédiateté ! Mais la justice des mineurs, ce n’est pas cela, ce ne peut pas être cela ! Enfin, nous saluons la suppression de l’article 5, qui visait à encourager les juridictions à déroger au principe d’atténuation de la peine.

on dénombre environ 800 mineurs incarcérés chaque mois depuis 2024, contre 700 au cours des dernières années. Il n’y a pas non plus d’explosion de la délinquance chez les jeunes : la part des mineurs impliqués dans les délits commis est passée de 22 % en 1998 à 12 % en 2023. La commission a bien souligné, dans son

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous resterons attentifs à l’évolution de ce texte au cours de son examen, d’autant qu’un grand nombre d’amendements visant à rétablir des mesures problématiques y seront discutés. S’ils sont adoptés, nous nous opposerons à ce texte. Nous continuerons à défendre la spécificité de la justice des mineurs et à nous opposer à son rapprochement avec la justice des majeurs.

est aussi d’appréhender cette question avec un minimum de rigueur et de distanciation par rapport à l’émotion que provoquent ces drames. Pour cela, j’aimerais rappeler quelques éléments factuels. Selon les chiffres du ministère de la justice, en 2022, dans les affaires relatives à la délinquance des mineurs traitées par les parquets, 168 900 mineurs

que pour les majeurs : comme M. le garde des sceaux l’a souligné tout à l’heure, 816 mineurs étaient incarcérés le 1 octobre 2024, contre 214 en janvier 2023.

et qui permet d’acter la responsabilité, puis l’audience de sanction. Entre les deux, dans un temps contraint, a lieu une phase de mise en œuvre d’un travail éducatif, l’on pourrait presque qualifier de séquence de probation. Mes chers collègues, si nous supprimions ce processus,

des mineurs, à savoir l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge, la primauté de l’éducatif sur le répressif et la spécialisation de la justice des mineurs.

proscrite par le Conseil constitutionnel en 2011. Il inversait le principe de l’atténuation des peines pour les mineurs de plus de 16 ans, laquelle deviendrait l’exception, mesure soulevant aussi une question constitutionnelle au regard du principe de proportionnalité. Enfin, il aggravait les sanctions envers les parents. ce texte relevait plus de la réaction à l’actualité que de la volonté de corriger les faiblesses structurelles de la justice des mineurs, à savoir l’inapplication des peines prononcées par le juge,

euros d’amende ? Le problème n’est il pas ailleurs ? Plutôt que d’adopter des mesures contestables et potentiellement inconstitutionnelles, ne devrions nous pas nous concentrer sur l’exécution des peines et le renforcement de notre institution judiciaire ? On ne peut pas, à la fois, dire qu’il faut prioriser l’éducatif et ne faire que du répressif ! C’est pourquoi, sans être totalement en phase avec la philosophie générale du texte, nous avons souscrit aux modifications effectuées par la commission. chers collègues, nous sommes inquiets au regard des amendements déposés en vue de la séance et du débat que nous avons eu en commission

se revendiquer de l’opinion publique pour faire voter des mesures manifestement inconstitutionnelles, d’attendre que ces mesures soient légitimement censurées, puis d’accuser le Conseil constitutionnel de bloquer la « volonté des Français ». Comme si l’argument de la constitutionnalité n’était plus un argument,

Ce qui est irresponsable, en revanche, c’est d’entraîner le Parlement dans une forme de trumpisme législatif, où l’on fabrique des textes pour l’affichage et où l’on teste la solidité du Conseil constitutionnel, à charge pour lui de souffrir la vindicte de l’opinion. Le critiquer sera d’autant plus facile

Le texte issu de la commission a donc été amélioré juridiquement sur la forme,… Tant mieux ! … c’est incontestable, mais aussi substantiellement modifié sur le fond. En écoutant le rapporteur, je me suis dit : « La réponse est non, mais, au fait, quelle était la question ? quelle était la question ? » Non, il ne s’agit pas d’une loi de circonstance. Ah bon ? Au delà des multiples faits divers récents, intolérables et inacceptables, nul ne peut nier que la violence des mineurs délinquants est de plus en plus grave, de plus en plus précoce – certes, en volume, elle diminue – et de plus en plus organisée. Pis, elle n’épargne plus aucun territoire, qu’il soit urbain ou rural. Les mineurs âgés de 13 à 17 ans ne comptent que pour 6 % de la population, mais représentent 40 % des mis en cause dans les vols avec violence, et le nombre de mineurs mis en cause pour coups et blessures volontaires sur d’autres mineurs de moins de 15 ans a augmenté – écoutez bien, mes chers collègues ! – de 350 % depuis vingt ans. Les mineurs sont toujours plus impliqués, on l’a dit ici, dans les narcotrafics, dans les rixes mortelles entre bandes rivales ou dans la délinquance de rue. Refuser de voir cette réalité alarmante, par posture idéologique, revient à nier ce que les Français subissent subissent au quotidien, alors qu’ils nous demandent, dans leur très large majorité, un durcissement de notre politique pénale, comme le souhaitent avec constance et cohérence le garde des sceaux et le ministre de l’intérieur. Ce matin encore, Bruno Retailleau… Voilà ! … a plaidé pour réformer profondément la justice des mineurs. Favorable à de courtes peines de prison de quelques semaines, il a souhaité étendre la comparution immédiate aux mineurs délinquants et faire en sorte que l’excuse de minorité soit non plus la règle, mais l’exception. Oui, la justice pénale des mineurs obéit à des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La création en 2021 du code de la justice pénale des mineurs a été une réforme ambitieuse, certes nécessaire, mais aujourd’hui très insuffisante face à l’augmentation exponentielle de la violence. Dans le prolongement de cette réforme, nous devons donc amplifier nos efforts dans les domaines de la responsabilisation des parents et du traitement des délinquants multirécidivistes.

des articles supprimés et à renforcer les garanties procédurales. La délinquance des mineurs est un sujet de préoccupation essentiel pour les Français. Ils attendent de nous une position forte. Il serait dommage d’apporter avec ce texte une réponse purement technique, plutôt que d’assumer nos responsabilités politiques.

société, où l’autorité des parents était respectée, où l’école imposait ses règles et où la justice n’excusait pas systématiquement. Mais ouvrons les yeux

Aujourd’hui, nous faisons face à une explosion de la délinquance juvénile ultraviolente : des bandes qui terrorisent nos quartiers, des violences gratuites, des professeurs agressés, des pompiers caillassés et, surtout, une criminalité qui atteint des sommets dans certaines villes.

de narcotrafiquants, mais aussi par une armée de tueurs à gages mineurs. Oui, mes chers collègues, des adolescents de 14, 15 ou 16 ans exécutent pour quelques milliers d’euros. Ces gamins n’ont plus peur de rien, ni des balles adverses, ni de la police, ni des prisons, parce qu’ils savent que notre justice ne les sanctionnera jamais à la hauteur de leur crime. Il faut que cela cesse. À 16 ou 17 ans, on sait ce que l’on fait

que la République n’est pas une grande muette laxiste. Si certains adultes refusent d’éduquer leurs enfants, alors c’est au législateur de mettre la société à l’abri de ces bombes à retardement. Un jeune délinquant impuni devient un modèle de récidive, non de réhabilitation. Cessons donc de sacrifier la justice sur l’autel de la naïveté

Nous sommes collectivement responsables de ce sauvage assassinat, qui aurait dû être évité. Faute de moyens, mais aussi parce que nous n’avons pas fixé les bonnes règles, nous assistons, impuissants ou presque, aux ravages de l’hyperviolence juvénile. Il faut vraiment en finir avec cette culture de l’excuse, de l’impunité, du renoncement. Je salue l’initiative de Gabriel Attal, dont la proposition de loi comportait, en germe, des avancées significatives sur des thèmes que la majorité sénatoriale a toujours soutenus. C’est parce que nous avons aujourd’hui l’occasion d’inscrire nos convictions dans la loi que j’ai souhaité proposer la réécriture de certains articles supprimés et compléter cette proposition de loi en instaurant la possibilité d’ultracourtes peines de prison. Monsieur le garde des sceaux, il faut réévaluer en urgence la réforme qui a conduit à la césure du procès pénal des mineurs et en tirer les conséquences. La punition n’est pas l’antithèse de l’éducation, elle en est le corollaire. Je salue l’amendement de Lauriane Josende, dont les Attendre que le mineur s’enfonce dans la délinquance pour agir, c’est consacrer l’idée pernicieuse selon laquelle la justice, donc la société, recule face aux premières transgressions, les tolère, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. La première infraction doit être immédiatement sanctionnée, sans quoi nous organisons notre propre impuissance. Il est donc impératif de réintroduire la possibilité pour les juges de prononcer de très courtes peines d’emprisonnement. De telles peines sont une composante à part entière de l’éducation. Elles sont indispensables pour rappeler l’autorité de la loi et éviter la spirale de la récidive. Nous devons cesser d’invoquer la minorité comme un prétexte à l’inaction. Peut on sérieusement soutenir que des jeunes capables d’une violence extrême, d’une brutalité inouïe, doivent être jugés avec une indulgence quasi systématique, au seul prétexte de leur âge ? C’est Lorsque la gravité des faits l’exige, il est également décisif d’instituer la possibilité d’une comparution immédiate de mineurs déjà bien connus de la justice. Et pas de justice pénale à la carte : si le mineur ou ses parents refusent la comparution immédiate, le mineur doit pouvoir être placé en détention provisoire et être jugé dans les délais les plus brefs. Mes chers collègues, il nous appartient de rétablir l’autorité de la justice. Une justice beaucoup plus ferme et plus efficace, une justice qui protège les victimes et les mineurs eux mêmes. Il y va de l’avenir même de notre jeunesse. Car, ne l’oublions jamais, les premières victimes de cette hyperviolence juvénile, ce sont aussi et surtout des jeunes ! La parole

part, nous avons bien fait de venir… Nous ne sommes plus en 1912, date de parution du roman de Louis Pergaud, et Gérald Darmanin n’est pas le père Zéphirin, le garde champêtre de cet ouvrage. Les bandes qui s’affrontent aujourd’hui n’utilisent plus l’épée en bois ou la fronde, mais font régner la terreur à coups de machette, de couteau, de kalachnikov ou de chalumeau.

dans les failles du système, des mineurs délinquants deviennent des acteurs majeurs et récurrents de la galaxie mafieuse.

cette proposition de loi qui vise à lutter contre la délinquance des plus jeunes est pensée comme une réponse aux révoltes urbaines de l’été 2023. Mais, bien loin du désir de justice, vous menez un tout autre combat dans la continuité de la bulle populiste qui gangrène nos débats depuis des semaines, il nous est proposé d’examiner une loi établie sous le coup de l’émotion. C’est tout à fait contraire à ce que l’on attend du travail des parlementaires En écoutant les professionnels du secteur de la justice, ce que n’ont visiblement pas fait les auteurs de la proposition de loi, on se rend compte que nous sommes en présence d’un texte qui fédère contre lui. En partie désavoué en commission à l’Assemblée nationale, il a été complètement désavoué par la commission au Sénat. Ce texte conduirait la France à rompre avec ses engagements internationaux, notamment la Convention internationale des droits de l’enfant, selon la Défenseure des droits, mais aussi, parfois, à ne pas respecter les principes constitutionnels. vous appelez à raison au respect de l’autorité. Mais si, demain, l’autorité humilie, bien loin d’apaiser, elle ne fera qu’embraser la situation. Non contents de fragiliser des familles déjà éprouvées par des parcours complexes, vous vous mettez en porte à faux avec la réalité. En vous concentrant uniquement sur la réponse judiciaire et répressive, vous balayez d’un revers de main les avancées obtenues dans les domaines de la psychologie de l’enfant et de la justice des mineurs. Vous tournez le dos à ces faits et offrez, une fois encore, des gages à l’idéologie punitive. Les mesures d’accompagnement, d’assistance, de prise en main du mineur existent et donnent des résultats. Elles sont portées par des fonctionnaires, des éducateurs, des magistrats consacrant leur vie à ces jeunes qui, un jour, ont fait l’erreur de basculer. Il faudra dire à ces professionnels que le budget du ministère de la justice ne sera pas renforcé pour ce qui concerne la justice des mineurs ! À la place, vous proposez d’enfermer plus vite et plus longtemps… J’espère que vous garderez sur la conscience le fait que les jeunes, qui ont déjà un pied dans la criminalité, auront, grâce à vous, un pied dans le chômage, l’isolement social et la récidive !

au point de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants mineurs. Cet amendement tend donc, si cette soustraction a conduit leur enfant à commettre un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à condamnation, à les punir de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros

est à M. Joshua Hochart. Cet amendement vise à réintégrer l’alinéa 7, supprimé par la commission, afin de garantir une prise en compte plus juste des infractions commises par les mineurs dans l’aggravation des peines applicables aux parents défaillants. En limitant cette aggravation aux crimes et délits commis par le mineur, la commission a introduit, de fait, un joker juridique pour le parent défaillant, en excluant les contraventions du champ des infractions prises en compte. Or parmi celles ci figurent notamment les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours, qualifiées de contraventions de 5 classe. Pourtant, dans la réalité des infractions commises par les mineurs, de nombreuses atteintes aux personnes relèvent précisément de cette catégorie, tout comme les dégradations et les détériorations mineures. En ignorant ces faits, la commission crée une faille juridique qui affaiblit la portée du dispositif. Cet amendement tend donc à rétablir l’alinéa supprimé et à maintenir l’aggravation de la peine principale encourue pour le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales. Ainsi, la peine applicable serait portée à cinq ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende. L’amendement

Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches, qu’il s’agisse

terrorisent des commerçants, s’attaquent aux forces de l’ordre, à nos pompiers, et sèment le chaos en toute impunité. Il y a quelques années, nous pouvions encore parler de cas isolés ; aujourd’hui, nous faisons face à un problème de masse, à la banalisation de la violence, à une véritable perte de repères. Où sont les parents dans tout cela ? Quelle responsabilité portent ils dans les actes commis par leurs enfants ? La République ne peut plus fermer les yeux sur la réalité : une partie de ces mineurs évolue dans un cadre familial où l’autorité parentale est inexistante, que les parents soient totalement absents, démissionnaires ou complices. Notre amendement vise donc à frapper là où cela produit un véritable impact, en suspendant ou en supprimant les allocations familiales pour les parents d’enfants délinquants ou criminels. Mes chers collègues, nous vous demandons de voter en faveur de cet amendement, pour mettre fin au laxisme parental et rétablir une autorité plus que nécessaire aujourd’hui. C’est cela

ouvre droit seront versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’établissement qui accueille le mineur le temps du placement ». Cela signifie que, pendant ce temps, ce ne sont pas les parents ayant la charge de l’enfant qui reçoivent cet argent.

en cas de non présentation des parents à l’audience du juge statuant en matière pénale. Je le rappelle, en matière civile, le montant de la sanction

Afin d’impliquer davantage les parents dans la réparation d’un dommage causé par leur enfant mineur, et sans pour autant sanctionner indirectement les victimes de ce dommage, la commission des lois a amendé l’article 3

à revenir sur ce principe, le présent amendement vise à éviter que la participation des parents à l’indemnisation d’un dommage causé à l’occasion de la commission d’une infraction pénale par leur enfant mineur ne soit utilisée comme argument commercial, dans un contexte concurrentiel. Ainsi, de façon très concrète, toute clause contractuelle par laquelle un assureur s’engagerait, par principe et sans évaluation au cas par cas, à ne pas réclamer auprès des parents le reste

tout de même instituer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs. L’amendement s’appuie sur un constat simple : les délais entre l’infraction et le jugement sont trop longs, ils affaiblissent la portée pédagogique et dissuasive de la sanction. Cela compromet l’autorité de la justice et empêche de répondre à l’attente légitime des victimes. La possibilité de prévoir la comparution immédiate du mineur renforcera l’efficacité de la justice pénale ; la réponse judiciaire sera plus lisible et rapide, et adaptée à la gravité des faits comme à la personnalité du mineur.

Le mineur sera jugé le jour même ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables. Il n’y aura pas de justice pénale à la carte : si le mineur ou ses parents s’opposent à la comparution immédiate, ce qui est leur droit, l’intéressé pourra être envoyé en détention provisoire ou soumis à une mesure de sûreté, et il sera jugé dans des délais les plus brefs.

Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il s’agit d’instaurer une nouvelle procédure de comparution immédiate à audience unique, afin de garantir une réponse pénale plus rapide et mieux adaptée. Ce dispositif, strictement encadré, ne concernera que les mineurs de plus de 16 ans déjà condamnés pour des infractions graves passibles de plus de sept ans de prison et en état de récidive Il s’agirait donc d’une procédure exceptionnelle, réservée aux situations où le trouble à l’ordre public exige une réaction immédiate. Les mineurs pourront alors être déférés le jour même, ce qui garantira une justice plus efficace et plus lisible pour nos concitoyens.

le fait de] jeunes gens de quinze à vingt ans – qui terrorisent la capitale. Et, en face de cette armée encouragée au mal par la faiblesse des lois répressives et l’indulgence inouïe des tribunaux, que voyons nous ? Maintes causes ont aidé au pullulement de cette redoutable [délinquance] : […] la suppression quasi radicale de l’apprentissage qui jette à la rue les gamins de 13 à 20 ans alors qu’ils devraient [travailler], […] l’insuffisance des moyens de répression qui semblent s’affaiblir au fur et à mesure que grandit l’audace des [délinquants] et surtout ce fâcheux esprit de sensiblerie humanitaire. J’ai montré […] avec quelle indulgence les parquets en usent vis à vis des rôdeurs. On les relâche aussitôt arrêtés ou bien on les condamne à des peines minimes alors que, le plus souvent, ils auraient mérité pour le moins les travaux forcés. On abuse et on mésuse des lois de pardon et de sursis, de la libération conditionnelle, de la réduction des peines. Et, quand on ne peut faire autrement que [de condamner] et d’envoyer les délinquants en prison, c’est dans des prisons confortables qu’on les loge, dans des prisons où ils trouvent bon gîte et bon repas, de l’air pur, des livres pour se distraire et si peu de travail à faire que ce n’est pas la peine d’en parler. » Ce texte provient du du 20 octobre 1907.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

Toutefois, force est de constater que cette faculté est étroitement encadrée et peu utilisée par les parquets. L’amendement vise à faciliter le recours à la procédure d’audience unique en abaissant le quantum de peine d’emprisonnement encourue à compter duquel un mineur peut être jugé sans césure sur l’initiative du parquet : trois ans pour les 13 16 ans et un an pour les mineurs de plus de 16 ans. Mes chers collègues, en votant cet amendement, vous contribuerez grandement au renforcement de notre arsenal juridique en améliorant la qualité de notre réponse pénale. Quel